aux voix. Je mets aux voix le texte adopté par la commission sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Moldavie relatif à l'emploi salarié des conjoints des agents des missions officielles de chaque État dans l'autre, de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Bénin relatif à l'emploi salarié des personnes à charge des agents des missions officielles de chaque État dans l'autre, de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Serbie relatif à l'exercice d'une activité rémunérée des membres des familles des agents des missions officielles de chaque État dans l'autre et de l'accord entre le gouvernement de la République française et le conseil des ministres de la République d'Albanie

D'une part, la multiplicité des usages offerts par ces données permettra la mise en place d'innovations dans notre processus de construction et se traduira par un gain qualitatif pour les pour les futurs occupants des logements. D'autre part, cette mesure s'inscrit dans la démarche d'efficacité et de simplification qui anime le projet de loi. L'accès à des données représente en effet de nombreuses opportunités pour permettre un gain de temps considérable dans le processus de construction. Je tiens à préciser que cette disposition ne présente aucun risque pour la vie privée des propriétaires et qu'elle respecte les dispositions du règlement européen sur la protection des données personnelles. Les informations respecteront les exigences d'anonymisation. En d'autres termes, les données disponibles ne permettront en aucun cas d'identifier les propriétaires et seront garantes vis-à-vis du secret fiscal. Vous l'avez compris, cet amendement, qui avait reçu un double avis favorable à l'Assemblée nationale, va dans le sens de la simplification,

cet article. Contrairement à ce que vous venez de soutenir, monsieur Patriat, nous avons pensé que les données qu'il est prévu ici de rendre publiques sont couvertes par le secret fiscal et qu'elles ne sauraient être divulguées sans ciblage particulier ni véritable garantie d'anonymisation.

et l'anonymisation des données nécessiteraient des travaux informatiques incompatibles avec les opérations prioritaires de refonte de l'application MAJIC

prévoit dans sa rédaction actuelle que le projet d'aménagement et de développement durable, le PADD, fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain en lien avec l'analyse de la consommation passée. La commission des affaires économiques complète cet article pour préciser que ces objectifs tiennent compte de la taille des parcelles des communes de montagne ou des communes de faible densité démographique. Il convient de rappeler que, contrairement à ce qui était indiqué dans l'exposé des motifs de l'amendement adopté en commission, ces dispositions n'ont pas été votées par le Sénat dans la rédaction proposée, au motif qu'elles étaient insuffisamment précises. Par ailleurs, l'analyse du potentiel de densification permet de prendre en compte les spécificités de tous les territoires, y compris les espaces très ruraux. Je vous propose donc de supprimer cet article, mes chers collègues. Quel est l'avis de la commission ? Il sera

les objectifs fixés par le PADD. Ce dernier doit justement refléter les réalités du territoire et tenir compte de ses spécificités. La taille des parcelles doit donc être prise en compte dans l'établissement des objectifs. Quel est l'avis

Plutôt que d'étendre le champ des exceptions à l'infini, une réflexion aurait pu être menée avec tous les acteurs du secteur pour actualiser ce texte et tenir compte de différentes évolutions.

qui régiraient désormais les relations entre certains maîtres d'ouvrage publics et les maîtres d'oeuvre, et ce afin de compenser l'affaiblissement des dispositions de la loi MOP. Sans cela, le projet de loi laisserait un vide dangereux qui, j'insiste sur ce point, fait craindre, et pas seulement aux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 proposons qu'un décret en Conseil d'État vienne préciser les conditions d'application de l'article 3 de la loi de 1977, en particulier le contenu du contrat qui lie le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre, ainsi que le périmètre et les modalités d'intervention de l'architecte au cours de la réalisation de l'ouvrage. Notre objectif est également de mieux déterminer les responsabilités de chaque prestataire. Rappelons que le régime de responsabilité de chacun était clairement défini sous l'empire de la loi MOP. Eu égard aux multiples dérogations introduites par ce projet de loi, qu'en sera-t-il désormais ? D'ailleurs, nous constatons que l'étude d'impact est muette sur cette implication. En conséquence, le décret peut constituer une issue favorable pour apporter une véritable sécurité juridique, désirée par l'ensemble des prestataires. Ces derniers craignent, rien de moins, une augmentation sensible du contentieux en cas de difficulté ou d'erreur de construction Quand les responsabilités sont mal définies, ce sont des procédures judiciaires qui sont enclenchées et des retards qui s'accumulent, soit l'effet exactement inverse de celui qui est recherché avec ce texte. Quel est l'avis de la commission

Les maîtres d'ouvrage privés doivent être libres de définir le contrat et les missions qu'ils confient aux maîtres d'oeuvre privés en fonction de leurs besoins et des attendus du projet.

Afin de garantir aux usagers, mais aussi aux maîtres d'ouvrage, bailleurs sociaux ou promoteurs privés, la qualité des logements et la conformité de leur réalisation, que ce soit dans le cadre d'une construction neuve ou d'une rénovation, il est nécessaire, conformément à l'article 3 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture, de permettre à l'architecte de contrôler les études d'exécution et la réalisation des travaux tout au long du processus de construction.

Les compagnies d'assurance font d'ailleurs le lien entre la baisse de sinistralité et la présence de l'architecte sur le chantier. Cette mission s'inspire de celle qui a été adoptée à l'article 91 de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine concernant l'identification de la maîtrise d'oeuvre dans les marchés publics globaux. La parole pour présenter l'amendement n° 685 rectifié. L'esprit de ce projet de loi est de desserrer un encadrement tatillon du secteur de la construction en termes de normes imposées, et donc de coûts et de délais. cet objectif et je pense qu'il est sain de remettre un peu de bon sens dans tout cela. Pour autant, il faut faire très attention à la qualité des bâtiments qui émergeront de ces constructions. Il faut peut-être construire vite, mais pas n'importe comment. Cet amendement s'inspire de l'expérience bordelaise de l'opération d'intérêt national Bordeaux-Euratlantique et ne vise, bien évidemment, que les logements collectifs. Le fait que l'architecte suive les différentes étapes des travaux me paraît constituer un gage de sérieux, et

Aujourd'hui, cela dépend de la volonté du maître d'ouvrage. Cette mission constituerait une garantie supplémentaire de la qualité du bâti et elle protègerait non seulement le maître d'ouvrage, mais également les destinataires des bâtiments. Nous estimons qu'il est nécessaire, conformément à l'article 3 de la loi de 1977 sur l'architecture, de permettre à l'architecte de contrôler la construction du bout en bout les études d'exécution jusqu'à la réalisation des travaux et tout au long du processus de construction. Il s'agit, au fond, comme pour un pâtissier, de permettre à celui qui a fait la recette de la préparer.

et la cohérence des travaux avec le permis de construire jusqu'à la délivrance de la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux. Il n'est pas anodin que les compagnies d'assurance fassent le lien entre la baisse de sinistralité et la présence de l'architecte sur le chantier. L'architecte, de par sa place, n'est pas soumis aux impératifs financiers. Il est le garant de la bonne construction selon ses plans de réalisation. Cette mission s'inspire de celle qui a été adoptée à l'article 91 de la loi dite « LCAP » concernant l'identification de la maîtrise d'oeuvre dans les marchés publics globaux.

Cette mission n'a vocation à s'appliquer que dans le cadre de la réalisation de logements collectifs ou de groupements d'habitations de plus de deux logements. Elle ne s'appliquera donc pas aux particuliers. Quel

en particulier aux cages d'escalier de service, aux puits de lumière ou aux courettes, qui avec le temps et l'usage ont perdu de leurs fonctions initiales et ne sont finalement plus que des zones de déperdition énergétique. amendement vise à indiquer que le règlement du plan local d'urbanisme peut fixer des règles permettant l'extension des parties privatives sur de telles parties communes, conformément à la décision de l'assemblée générale des copropriétaires, afin d'optimiser l'utilisation des surfaces et d'améliorer les performances énergétiques des constructions.

Vous l'aurez compris, nous avons entendu la colère des associations représentant les personnes en situation de handicap, qui qualifient cette mesure de grave régression. Nous partageons avec elles cette indignation légitime. Vous me direz, ce n'est pas le premier recul en la matière, mais quand même vous touchez à un totem, celui de la société inclusive, celui de l'ambition pour notre société de ne pas laisser sur le bord du chemin une partie de la population. Vous touchez à l'exigence de solidarité. Je ne suis pas sûre que le compromis trouvé en commission saura convaincre. Il reste pour nous inacceptable. La dernière enquête de l'INSEE est claire. Seuls 40 des 350 000 appartements et maisons individuelles, tous statuts d'occupation confondus, construits chaque année entre 2006 et 2014 répondent aux règles d'accessibilité et d'adaptabilité fixées par la loi Handicap de 2005 et l'ordonnance du 26 septembre 2014. C'est extrêmement peu. Ce n'est donc le moment ni de renoncer, sous couvert d'économies, à ce principe fort d'accessibilité ni de renforcer les inégalités. le Gouvernement nous fait la démonstration qu'il se montre dur avec les faibles et faible avec les forts. J'entends déjà les cris de joie des promoteurs à l'idée de faire quelques mesquines économies sur le dos des personnes en situation de handicap. quelques mètres carrés en moins pour les habitations : jamais, en effet, vous ne nous ferez croire que les quelques mètres carrés grappillés dans les entrées et les salles de bains seront ventilés ailleurs.

Vous appliquez la double peine pour ces personnes qui cumuleront handicap et difficultés d'accès au logement. J'ajoute que cette situation est aussi en parfaite contradiction avec les ambitions de la loi sur l'adaptation de la société au vieillissement, qui

contrairement au texte initial, qui prévoyait un seuil de 10 %. Cette mesure va malgré tout à l'encontre des besoins quantitatifs et qualitatifs des personnes handicapées et âgées ; elle constitue une grave régression sociale. On passerait ainsi de 100 % de logements neufs accessibles, comme le prévoyait la loi Handicap de 2005, à la notion floue et indéfinie de « 100 % de logements évolutifs », autrement dit de logements susceptibles d'être adaptés pour accueillir une personne handicapée. Mais du coût des modifications ? ? du locataire qui n'aura plus la capacité de modifier son logement, voire de recevoir et d'accueillir des personnes handicapées ? Le Conseil national consultatif des personnes handicapées, le CNCPH, la Confédération nationale du logement et l'Association nationale pour l'intégration des personnes handicapées moteur, l'ANPIHM, ont publiquement dénoncé cette « très forte réduction des normes d'accessibilité dans la construction de logements neufs », et un collectif de treize organisations représentatives des personnes en situation de handicap et de la lutte contre l'exclusion a fait part de sa parfaite incompréhension face à ces mesures « en incohérence totale avec les autres politiques publiques engagées par le Gouvernement, ainsi qu'avec le vieillissement de la population Il est important de souligner que le quota proposé dans ce texte ne porte pas sur 100 % des logements nouveaux, mais sur 100 % des logements nouveaux réputés accessibles les parties communes, c'est-à-dire, notamment, ceux qui sont desservis par un ascenseur ou situés en rez-de-chaussée. Selon les calculs de l'ANPIHM, sur les 45 000 logements HLM construits chaque année, seuls 23 000 peuvent accueillir une personne en fauteuil roulant avec l'application du quota de 30 %, ce chiffre tomberait à 6 900, et il serait de 2 300 pour un quota de 10 %. Il n'y aurait donc plus qu'un appartement HLM accessible supplémentaire par tranche de 32 000 habitants. Il ne s'agit là que des seuls logements sociaux ; dans le secteur privé, le constat sera bien pire. Je considère que l'instauration d'une politique de quotas conduira à la réduction drastique d'une offre déjà très insuffisante de logements immédiatement habitables sans travaux, d'où la nécessité d'une suppression de l'article 18.

Un quota de 30 % plongera les personnes handicapées dans la précarité sociale et compromettra leur accès au logement. Cela les contraindra à revoir leurs critères au rabais afin de pouvoir se loger, ou à choisir leurs relations sociales selon des critères d'accessibilité.

Ce texte de régression sociale contredit les objectifs d'autres politiques publiques engagées par le Gouvernement, notamment le développement de l'habitat inclusif et de l'hospitalisation à domicile, ainsi que l'élévation du handicap au rang de priorité du quinquennat en 2017. De plus, il viole les engagements internationaux auxquels la France a souscrit, notamment l'article 19 de la convention relative aux droits des personnes handicapées de l'ONU, ainsi que la résolution du Conseil de l'Europe du 15 février 2001, selon laquelle « la conception universelle et l'accessibilité ont un rôle de premier plan à jouer dans la promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». Cet article 18 met tout simplement en place une revendication de longue date du du bâtiment et, en particulier, de la Fédération française du bâtiment, qui réclamait mot pour mot une telle mesure dès 2013. Il est le reflet du désengagement de l'État face aux questions sociales. Il vise en effet, purement et simplement, à diminuer les coûts de construction au bénéfice des propriétaires, et ce bien que les coûts induits par les fluctuations des marges commerciales-

mes chers collègues, sur les enjeux de cette simplification outre-mer. Vous n'ignorez pas que le secteur de la construction est crucial pour le bien-être économique et social de nos territoires, où nous sommes confrontés à d'immenses besoins en logements et aménagements structurants, qu'à des défis colossaux résultant de contraintes multiples : surcoûts liés à l'éloignement et à l'étroitesse des marchés locaux, exiguïté du foncier disponible, climats particulièrement corrosifs et exposition accentuée aux risques naturels. À ces nombreuses contraintes viennent s'ajouter le poids des normes et leur fréquente inadaptation aux réalités ultramarines. C'est pourquoi la délégation sénatoriale aux outre-mer a choisi, en 2017, de se plonger dans la nébuleuse normative pour aboutir à une trentaine de propositions visant à faire cesser les anomalies paralysantes et autres situations ubuesques, mais également à valoriser les ressources locales et les démarches innovantes. À ce titre, je défendrai plusieurs amendements, inspirés de nos travaux, tendant à mieux prendre en compte les spécificités ultramarines dans la production des normes et à mieux mesurer les surcoûts d'assurances. c'est en desserrant l'étau normatif que nous parviendrons outre-mer à simplifier l'acte de construire. Alors, je vous demanderai, mes chers collègues, de considérer que, derrière chaque amendement que je présente, il n'est jamais question de précisions superflues, mais d'une réelle volonté de changement : les normes produites doivent prendre en compte les latitudes sous lesquelles elles s'exercent ! Enfin, permettez-moi un dernier mot pour regretter que que la commission ait jugé irrecevable, au titre de l'article 45 de la Constitution, un amendement que j'avais déposé. Son objet était d'expérimenter, à Mayotte et en Guyane, une simplification des constructions scolaires, en permettant aux communes de déroger à certaines règles en vigueur en matière de marchés publics. Là encore, il ne s'agissait pas de déroger pour déroger, mais de répondre à une réalité : en raison de procédures souvent longues et coûteuses, les élus sont aujourd'hui dans l'incapacité d'anticiper les effectifs.

C'est la raison pour laquelle, au vu de toutes ces contraintes, le précédent gouvernement et, notamment, Mme Ségolène Neuville sont revenus sur un certain nombre de mesures à la demande de l'Association des maires de France, de l'Association des maires des petites villes de France et de l'Association des maires ruraux de France. On pouvait en effet pour la mise en accessibilité des logements, des mairies et des services publics étaient intenables et n'étaient absolument pas finançables. Il ne s'agit pas de donner de l'argent aux plus riches ou aux promoteurs, mais de permettre aux collectivités locales et à nos offices d'HLM de s'en sortir.

Ce positionnement est incohérent avec la volonté annoncée du Gouvernement de modifier l'offre médico-sociale et de tendre vers une société plus inclusive, ce qui demande, de fait, un nombre de logements plus important. Ce quota de 10 %, qui ne concerne que les logements accessibles par ascenseur ou situés en rez-de-chaussée, est en deçà des besoins de la population touchée par le handicap, dont la proportion est estimée à 15 %. Rappelons que plus de 20 % des Français auront plus de soixante-cinq ans en 2025. L'accessibilité concerne également les personnes en perte d'autonomie. De plus, cette disposition est contraire au principe d'accessibilité universelle, principe général repris par tous les gouvernements. De nombreuses questions restent en suspens, monsieur le ministre. Quelle est la définition d'un logement évolutif ? Quel est le délai raisonnable pour adapter un logement ? Qui finance les travaux de mise en accessibilité ? Je souhaiterais vous entendre sur ces points. Je tiens à saluer le travail de la commission des affaires économiques et de Mme le rapporteur, qui ont fait évoluer le texte en proposant deux mesures visant, l'une, à augmenter le nombre de logements qui devront être accessibles, dans les bâtiments d'habitation collectifs neufs, en portant le taux à 30 et l'autre, importante, à modifier les critères prioritaires d'accès au logement en faveur des personnes handicapées, de façon à ce que les logements accessibles soient bien destinés aux personnes qui en ont besoin. Ces deux mesures parallèles sont essentielles. J'espère que cette solution de compromis, quoiqu'imparfaite au regard du principe d'accessibilité universelle, permettra tout de même de mieux répondre aux besoins des personnes en situation de handicap qui, rappelons-le, disposent souvent de revenus modestes et vivent parfois dans un isolement social intolérable. La parole

inquiétude peut-être légitime ; néanmoins, la caricature et les faux problèmes ne peuvent pas être retenus. Quant à nous, notre rôle, en soutien au Gouvernement, est d'entendre ces craintes et d'y répondre.

n'est pas une science exacte et nous avons raisonné ainsi : si l'on applique cette proportion au parc de logement existant en France, soit 34 millions de logements, un quota de 10 % correspondrait environ à 3,5 millions de logements accessibles ; pour 850 000 personnes à mobilité réduite, cela nous semble raisonnable.

Elle espère que le Sénat ne va pas abaisser la norme d'accessibilité issue de la loi du 11 février 2005. « C'est une question d'égalité et de dignité, déclare-t-elle, et cela permettrait au législateur de signifier clairement que l'inclusion des personnes en situation de handicap lui importe. » Oui, cette question nous importe, monsieur le ministre ! L'accessibilité ne peut pas être réduite à des considérations techniques. Je tiens à saluer la démarche de Mme la rapporteur, qui a essayé de trouver un compromis avec le Gouvernement, mais l'accessibilité ne peut pas faire l'objet de solutions de compromis, car elle conditionne la concrétisation des droits des personnes handicapées et elle est un préalable nécessaire à leur participation sociale. S'il est un projet politique humaniste qui peut encore nous mobiliser, c'est bien celui de la construction d'une société plus inclusive, ouverte à tous et respectueuse des différences. L'accessibilité en est un des principes fondateurs. Le projet de loi ÉLAN ne constitue pas seulement un recul du droit au logement pour les personnes en situation de handicap et une remise en question des engagements internationaux de la France ; il est porteur d'exclusion et de discrimination, et révèle combien le Gouvernement ignore ces enjeux de société qui ont vocation à améliorer la qualité de vie de tous.

de trois étages. Par cet amendement, nous entendions traduire législativement un engagement du Gouvernement. En effet, face à la colère des personnes handicapées contre la baisse du quota de logements accessibles prévue dans ce texte, le Gouvernement tenterait de rectifier quelque peu le tir. Un décret serait en préparation pour rendre obligatoire l'installation d'un ascenseur dans les logements neufs de trois étages. Nous avions ici l'occasion de transformer les promesses en une mesure législative en bonne et due forme. Aujourd'hui, selon le code de la construction et de l'habitation, les constructeurs ont l'obligation d'installer des ascenseurs dans les immeubles comptant quatre étages et plus. Cette restriction allège considérablement la portée de cette obligation. En effet, hors métropoles, les immeubles construits n'excèdent pas trois étages au-dessus du rez-de-chaussée. Cette situation est source d'une importante discrimination de fait pour les personnes en situation de handicap et utilisant des fauteuils roulants, ainsi que pour l'ensemble des personnes à mobilité réduite. Je rappelle que la France est l'un des seuls pays d'Europe, avec la Hongrie et la République Tchèque, à maintenir le seuil à quatre étages et plus. visait à instituer l'obligation d'installation d'un ascenseur à partir de trois étages. C'est d'ailleurs une revendication importante de l'Association nationale pour l'intégration des personnes handicapées moteur. Une enquête Ipsos menée en décembre 2017 révèle par ailleurs que 74 % des Français considèrent nécessaire d'installer un ascenseur dans les immeubles de moins de quatre étages, tandis que, pour 48 % des Français, la présence d'un ascenseur est un élément décisif pour choisir un logement. Nous souhaitions donc traduire législativement les engagements du Gouvernement.

défini ce qu'est un logement évolutif. C'est avec ces associations que nous sommes en train de finaliser les normes et les décrets qui

avons tout à fait répondu, monsieur le sénateur. Il y a deux possibilités. Vous avez les logements sociaux et les logements dits « privés ». Dans les logements sociaux, les bailleurs

contre 100 % aujourd'hui, en remplaçant cette obligation de construire des habitations accessibles par celle de bâtir des logements évolutifs. Cette disposition, outre le fait qu'elle est floue sur ses financements et son application, est de nature discriminante et inégalitaire. Par sa volonté affichée de simplifier les normes de construction, le projet de loi condamne les personnes handicapées à ne plus pouvoir choisir librement leur lieu de vie, ce qui est en totale contradiction avec l'article 19 de la convention de l'ONU relative au droit des personnes handicapées. Faut-il rappeler que cette De nombreuses organisations représentatives des personnes en situation de handicap ont exprimé leur surprise et leurs inquiétudes face à cette régression qui bafoue les droits des personnes handicapées inscrits dans la loi de 2005, si chère à l'ancien sénateur Paul Blanc. Ce dispositif est aussi en contradiction avec les autres politiques publiques actuelles qui visent à rendre la société plus inclusive. Enfin, il va à l'encontre des adaptations nécessaires à l'évolution de notre population, qui comptera une personne sur trois âgée de soixante ans et plus en 2050. Je rappelle que le Défenseur des droits, M. Jacques Toubon, a condamné de la façon la plus ferme cet article 18. Le Conseil national consultatif des personnes handicapées s'y oppose lui aussi. La Commission nationale consultative des droits de l'homme a dénoncé le principe même des 90 % de logements évolutifs, donc des quotas. Le Conseil de l'Europe, quant à lui, vient d'épingler et de mettre en garde la France, le vendredi 13 juillet dernier, sur la création de quotas de logements accessibles. Pour l'ensemble de ces raisons, nous souhaitons la suppression de cet article,

pour objectif de renforcer le maintien à domicile et le développement de l'ambulatoire, avec de plus en plus de soins dits de suite qui se font

revient ainsi sur une loi socle de notre République : la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, qui prévoit que l'intérieur et l'extérieur des locaux d'habitation sont accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap. L'article 18 va également à l'encontre de la nécessité de prendre en compte tant le handicap que le vieillissement de la population, à un moment où le Gouvernement lui-même promet des mesures en ce domaine. entre cet article et le maintien à domicile des personnes âgées défendu par la ministre de la santé ? Rappelons que près de 5 millions de Français auront plus de ans en 2050. La France a pris beaucoup de retard en matière d'accessibilité. Or, comme l'a relevé le Défenseur des droits dans un avis du 11 mai 2018, il faut appréhender l'accessibilité comme un véritable enjeu de notre société et anticiper les conséquences sociales et économiques de l'allongement de l'espérance de vie et de l'augmentation du nombre de personnes âgées en perte d'autonomie.

le propriétaire privé qui va accepter d'engager des travaux, et donc des frais, pour procéder à l'adaptation d'un logement afin de le louer à une personne en situation de handicap ? Cette mesure risque d'entraîner une discrimination supplémentaire pour l'accès au logement des personnes handicapées.

Contrairement à ce que dit le Gouvernement, c'est totalement insuffisant pour répondre aux besoins des 850 000 personnes en situation de handicap et cela ne répond absolument pas aux besoins futurs de notre population, à son vieillissement, et à l'augmentation du nombre de personnes âgées en perte d'autonomie. Notre groupe demande donc la suppression de l'article 18. Quel est

Didier Guillaume a dit que Jacques Chirac avait fait une bonne loi. Un Corrézien ! Il a raison, mais si on lui indiquait que les logements peuvent être évolutifs, je ne pense pas qu'il serait contre.

qui aura des coûts fatalement supérieurs à ceux que l'on aurait eu à supporter au moment de la construction initiale. Vous le savez très bien. Quelle est la cohérence entre l'annonce de votre société inclusive et la raréfaction de l'offre de logements accessibles ? Aucune ! Pas de cohérence, pas de rentabilité et, à mon sens, pas non plus la sacro-sainte efficacité que vous revendiquez tous les jours Peut-être aurait-il mieux valu se pencher sur la question de l'accessibilité universelle au moindre coût. Ainsi, nous aurions eu le mérite de ne pas contrevenir aux droits des personnes en situation de handicap, de respecter le principe républicain de l'égalité ... de préparer l'avenir, qui, comme vous le savez, puisque vous le dites souvent, ne doit jamais être insulté. C'est pourtant exactement ce que vous faites avec cette mesure.

S'il était adopté en l'état, ce projet de loi conduirait à une diminution significative de la proportion de logements accessibles aux personnes en situation de handicap que les bâtiments d'habitation collectifs neufs doivent obligatoirement J'espère que le Sénat français n'abaissera pas la norme en vigueur, telle qu'elle résulte de la loi de 2005. C'est une question d'égalité et de dignité, et cela permettrait au législateur de signifier clairement que l'inclusion des personnes en situation de handicap lui importe.

nous sommes dans une société qui ne permet plus ce qu'on appelait le parcours résidentiel. Aujourd'hui, une famille qui entre dans un logement social, dans certaines grandes villes de France, et même dans des zones un peu moins peuplées, n'a plus guère d'espoir

les élus, mais aussi les propriétaires privés et les bailleurs publics sociaux. Il nous faut trouver des solutions. On peut comprendre les inquiétudes des organisations représentatives des personnes en situation de handicap, du Conseil national consultatif

influents. Comment aborder ces sujets sensibles sans pénaliser les personnes en situation de handicap et de dépendance ?

Travaillons avec eux pour qu'ils fassent en sorte que ces mètres carrés soient mieux utilisés ! On a eu deux ou trois occasions de montrer qu'on pouvait mettre aux normes des logements d'une façon différente

vote. Je suis sensible à l'argument de l'adaptabilité et de l'évolution des logements. C'est un problème majeur. Cela a été dit, au cours de la vie, les situations changent et même

Cela étant, je retire mon amendement au profit de la proposition de la commission, qui vise à porter le seuil à 30 %. Je forme le voeu, messieurs les ministres, qu'elle s'applique à tous et sur tout le territoire.

le maintien à domicile de nos personnes âgées dépendantes. Comment faire en sorte que ces ambitions se conjuguent si nous n'avons pas mis en place les conditions pour que, dès le départ, au moins 30 % des logements concernés soient accessibles ? Par ailleurs, et j'y reviendrai au travers d'un amendement que nous défendrons, qu'est-ce

La parole est à M. Pascal Savoldelli,

nous apprêtons à acter en renonçant aux 100 %, se fait au bénéfice d'un dispositif, qui, en fait, sur le plan réglementaire, va être très complexe,

de 8 millions de nos concitoyens sont en situation de suroccupation. Les dispositions que nous portons visent justement à redonner des mètres carrés utiles, dès lors que cela est possible.